À quinze heures, le soir et la nuit : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

La refonte de cet article, rendue nécessaire par l'avis sévère du Conseil d'État, qui a pointé un risque majeur d'inconstitutionnalité, permet notamment d'éviter une double incrimination pour les mêmes faits et une rupture d'égalité devant la loi pénale. rédaction accroît la lisibilité et la clarté des nouveaux délits prévus, avec une délimitation claire et dénuée d'ambiguïté, fondée sur l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction. Plutôt que de conserver des dispositions différentes selon les milieux, nous avons également fait le choix d'un champ infractionnel visant à la fois les sols, l'air et l'eau, pour pouvoir mieux prendre en compte les pollutions aquatiques, atmosphériques et pédologiques. La commission a en outre fait le choix de ramener à sept ans la durée minimale permettant de définir la notion d'effets nuisibles durables. Nous avons enfin supprimé le terme d'écocide, qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle pouvant être reconnue à l'échelle internationale. Ce serait source de confusion d'introduire en droit interne

Comme nous pouvons le constater chaque jour, en ouvrant le journal, en allumant notre télé ou notre radio, la criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l'échelle internationale. Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché d'activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites rares. Quand elles existent, les sanctions sont particulièrement légères. En dépit de la particulière particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur caractère intentionnel et des dommages irréversibles qu'ils peuvent entraîner sur les écosystèmes et les conditions mêmes d'existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante. Les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d'un droit pénal de l'environnement qui permette de lutter vraiment contre les crimes qui menacent la planète. Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d'introduire dans notre arsenal juridique l'incrimination l'incrimination d'écocide par destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème. On désigne ici les crimes les plus graves, qui portent atteinte à la sécurité de la planète, pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty, juriste, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l'air, de l'atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore ou de leurs fonctions écologiques. Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l'écocide. Le choix du Gouvernement d'un délit

Cette mesure constituerait en effet le seul moyen efficace de prévenir les dommages graves, étendus et durables à l'environnement. Force est de constater que le Président de la République n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris à l'endroit de la Convention citoyenne. Non seulement la version du texte présentée par le Gouvernement ne reprend pas la définition du crime d'écocide proposée par les citoyens et citoyennes, mais, de surcroît, son délit d'écocide n'est en réalité qu'un délit de pollution. Nous réfutons cette vision court-termiste promue par certains grands groupes industriels, qui qualifient le crime d'écocide de frein à l'économie. Nous constatons, avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, les préjudices économiques, sociaux et environnementaux des actes perpétrés contre la nature et demandons une transition plus écologique et plus durable de nos modèles économiques. Le chlordécone a mis les filières essentielles de l'agriculture et de la pêche en péril d'une manière irrémédiable et, avec elles, la vie de milliers de femmes et d'hommes. C'est pourquoi la rédaction que nous proposons entend également faire entrer dans le champ du crime d'écocide la notion d'impact sanitaire, afin que puissent être prises en compte,

Il faut aller plus loin en termes de sanctions pour dissuader les contrevenants et protéger nos écosystèmes de la dégradation et de la destruction. Cet amendement tend donc à introduire dans notre loi pénale le crime d'écocide. J'ai déjà évoqué précédemment la nécessité de consacrer

Il ne faut donc pas craindre une répression généralisée en cas d'instauration d'un crime d'écocide. Le quantum des peines reflète par ailleurs la gravité du dommage causé à l'environnement. Les catastrophes environnementales qu'on a pu connaître ces dernières années ont eu des conséquences dramatiques, tant sur la nature que sur les populations. Il est normal, au regard des séquelles observées des années après, que les peines soient à la hauteur du préjudice subi par la nature. Enfin, pour compléter le dispositif, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le délit d'atteinte grave à l'environnement, pendant délictuel

Le Sénat a déjà rejeté, en mai 2019, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide. Le rapport de notre collègue Marie Mercier, au nom de la commission des lois, avait démontré de manière convaincante

n° 1471 serait incriminé « le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre,

Or le terme d'écosystème n'est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. Il s'applique donc à des échelles très différentes. Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve un étang pourrait ainsi se voir condamné pour un tel crime s'il choisissait de le détruire. Une telle incrimination est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, en raison de la disproportion manifeste entre le comportement réprimé et la peine encourue. Par ailleurs, cette nouvelle incrimination ne contiendrait aucune référence à la réglementation applicable en matière de protection

puisque serait réprimé le fait de causer des dommages graves à l'environnement, mais également le fait de causer des dommages de nature à mettre en danger la conservation des écosystèmes. La coexistence de ces deux conditions semble peu compréhensible. Je rappelle que le projet porté par le Gouvernement permet d'augmenter significativement la répression des atteintes graves à l'environnement,

toute une société de s'engager sur la voie d'un développement propre et durable ancré dans son environnement géographique direct. Notre groupe estimait opportun de mettre en place un mécanisme d'indemnisation des victimes de crimes environnementaux,

au motif qu'il aggravait une charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution, alors même que nous l'avions gagé. Il s'agit là d'une occasion manquée d'accorder enfin à ces victimes le moyen d'obtenir réparation de leur préjudice. Nous renouvellerons cette initiative

De nombreuses victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d'écocide. Il n'en sera rien. Après avoir enterré la demande de la Convention citoyenne pour le climat en intégrant une sorte de délit généralisé, et non un un crime, le Gouvernement et sa majorité ont créé un dispositif qui suscitera des débats juridiques sans fin. Le souhait de la Convention citoyenne pour le climat était pourtant de légiférer pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de ne garantir rien moins que l'habitabilité de la planète et, si possible, partout sur Terre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière aux auteurs des déprédations et en évitant d'abandonner à leur triste sort des populations entières vivant sur des territoires pollués. Avec la rédaction actuelle, je crains fort que les nombreuses victimes du chlordécone dans nos beaux départements de Guadeloupe et de Martinique n'obtiennent ni justice ni réparation. Vous faites en sorte que la loi de notre pays en reste à un simple délit. La France s'honorerait pourtant de ne pas attendre que le changement juridique intervienne au niveau international pour avancer sur cette question.

Le parc national des Calanques a été souillé par les boues rouges, et nous nous souvenons tous du littoral atlantique pollué par la dernière marée noire après le naufrage de l'en 1999. Doit-on s'en tenir à l'arsenal juridique que nous possédons actuellement ? Nous proposerons de nouveau d'inscrire le crime d'écocide dans ce texte, afin que la France puisse enfin poursuivre des faits qui sont aujourd'hui réprimés de manière presque anecdotique au regard de leur gravité. Les écocides sont certes rares, mais ils devraient être consacrés comme tels.

J'en citerai deux. Premièrement, les faits poursuivis doivent être subordonnés à la caractérisation du non-respect d'une mesure individuelle de l'administration, ce qui conditionne l'efficacité d'une telle mesure au renforcement des contrôles administratifs, seuls susceptibles de caractériser le non-respect de telles prescriptions. Or la mission d'information sur l'incendie de Lubrizol a révélé la diminution importante de ces contrôles durant les dix dernières années.

Ainsi, l'une des plus grandes catastrophes écologiques de ces trente dernières années n'entrerait pas dans la définition de ce nouveau délit. Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car possiblement contraire à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée, car inopérante. C'est pourquoi notre groupe propose de réécrire cet article pour répondre à l'objectif initial du projet de loi, à savoir créer une nouvelle infraction dans notre droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l'environnement, indépendamment de la réalisation d'un dommage ou d'une mise en demeure de l'autorité administrative.

tend ainsi à réprimer les comportements délibérés mettant gravement en danger l'environnement, et ce indépendamment de la réalisation d'un dommage ou d'une mise en demeure de l'autorité administrative.

Le présent amendement vise donc à transformer la circonstance aggravante de mise en danger de l'environnement en véritable délit de mise en danger de l'environnement. Nous ne serions cependant pas opposés à la possibilité de prévoir des peines moins élevées, comme nous l'avions proposé par le passé dans le cadre de l'examen d'autres textes. Tout d'abord, cet amendement vise à supprimer du caractère durable de l'infraction. Ensuite, il tend à sanctionner toute violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, ou un acte administratif individuel qui exposerait l'environnement à une dégradation substantielle. Il permet ainsi d'intégrer toutes les atteintes à l'environnement, y compris lorsque l'auteur méconnaît les dispositions d'autres codes que celui de l'environnement. Enfin, il a pour objet d'insérer ce nouveau délit au sein du code pénal, en cohérence avec l'article 410-1, qui reconnaît déjà l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation. Quel est

Il n'est pas souhaitable de créer pareil délit sans évaluation préalable ni étude d'impact. Il est nécessaire d'évaluer au préalable la manière dont cet article sera appliqué par les juridictions avant de créer un délit autonome. Quel est l'avis du Gouvernement ? Vous avez fait

ils visent à créer un délit autonome de mise en danger de l'environnement sans référence à la réglementation applicable à l'activité en cause. Nous préférons la rédaction de l'article 67 telle qu'adoptée à l'Assemblée nationale, qui circonscrit le champ d'application de la mise en danger de l'environnement et qui maintient l'équilibre de cette nouvelle incrimination.

pour faciliter le traitement des procès-verbaux. Nous créons de plus dans cet article 67 la circonstance aggravante du non-respect d'une mise en demeure en cas de mise en danger de l'environnement. Nous instaurons également un délit de pollution généralisée pour les pollutions les plus graves. Nous facilitons la reconnaissance de la récidive en matière de pollution, qui permet de doubler les peines, et nous mettons aussi en place

rendre le dispositif plus opérationnel. Cet article réprime les comportements qui font courir un danger grave à l'environnement, indépendamment de la réalisation du dommage.

Même dans le cas de dommages qui ont eu lieu, comme les conséquences des pollutions pour l'environnement sont très complexes à appréhender, il n'est que rarement possible de pouvoir montrer une telle durabilité.

qui emploie le terme « significatif » pour qualifier les atteintes à l'environnement. Le droit de l'environnement est déjà très complexe et difficilement appliqué sur le terrain- ce constat est partagé par tous. Cet article ne vient pas améliorer son efficacité,

Ce montant, qui m'apparaît plus dissuasif, permettra de réprimer plus efficacement ces comportements, qui créent un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement. Je rappelle que le non-respect d'une simple mise en demeure, sans mise en danger de l'environnement, est déjà passible d'une amende de 100 000 euros.

Le caractère durable des atteintes à l'environnement pourra être établi grâce au recours à des experts, comme cela est déjà le cas pour certaines infractions. Cet article a fait l'objet de nombreuses discussions avec l'ensemble des parties prenantes. Il aboutit à un équilibre

une atteinte est considérée comme durable : cette évolution répond en partie à la préoccupation des auteurs de cet amendement. En revanche, il me paraît nécessaire de conserver la notion d'atteinte grave, dans la mesure où il s'agit d'une circonstance aggravante en cas de non-respect de prescriptions administratives en matière d'installations présentant un danger pour l'environnement. Il est également nécessaire qu'un seuil, c'est-à-dire le nombre d'années à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, puisse définir la notion afin de limiter les divergences d'appréciation d'une juridiction à l'autre et de ne pas introduire de rupture d'égalité devant la loi pénale en fonction du lieu de commission de l'infraction.

et de diminuer en parallèle le montant de l'amende de 300 000 à 200 000 euros. Cet équilibre a paru plus conforme à l'objectif recherché, à savoir la volonté de réprimer la mise en danger de l'environnement de manière réaliste, dissuasive

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

ne pourra être sanctionné qu'après violation d'une autorisation administrative. Or les comportements de mise en danger de l'environnement, sans que le dommage se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d'une réaction administrative. administrative. Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l'environnement à l'ensemble des comportements régis par le code de l'environnement, même lorsqu'ils ne procèdent pas de la violation d'une prescription administrative. Dans sa rédaction actuelle, l'efficacité de cet article semble conditionnée au renforcement des contrôles administratifs- inspection des installations classées, police de l'eau ... Or la mission d'information sur l'incendie de Lubrizol

et réprimée par l'article du code pénal a pour fondement l'ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d'un acte administratif individuel.

que la prise d'un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer au moins dix années. L'évolution des connaissances scientifiques concernant le fonctionnement des écosystèmes rend cette appréciation par le juge particulièrement complexe »- on peut le comprendre ! Or j'entends souvent nos collègues de la commission des lois dire que la loi doit être précise et opérante.

Cependant, la rédaction actuelle pose problème. Elle crée simplement trois nouvelles incriminations sans qu'aucune des nombreuses infractions spéciales préexistantes soit remplacée. Cela a pour effet de complexifier davantage un édifice pénal déjà difficilement maîtrisable. De plus, comme pour l'article 67, la rédaction actuelle est inopérante du fait de l'utilisation du qualificatif « durable ». L'atmosphère et les milieux aquatiques étant deux environnements aux forts pouvoirs de dilution, il sera impossible de démontrer que les effets d'une atteinte à l'eau ou à l'air sont graves et durables, c'est-à-dire qu'ils perdurent au moins dix ans, comme l'exige pourtant le projet de loi. Enfin, la caractérisation du nouveau délit général d'atteinte aux milieux physiques nécessitera d'apporter la preuve d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, excluant les fautes d'imprudence et de négligence, pourtant les plus nombreuses. Cet amendement vise donc à créer des infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l'environnement, en créant un véritable délit d'atteinte à l'environnement, revenant à la rédaction initiale proposée en novembre 2020 par le garde des sceaux et la ministre de la transition écologique. L'amendement

au sein de différents codes, ainsi que d'une définition de l'infraction en fonction du non-respect d'une décision administrative. Cet éparpillement affaiblit la portée du droit pénal de l'environnement et sa vertu préventive. Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l'environnement et du développement durable et de

est trop souvent composée d'infractions d'une grande technicité exigeant la démonstration d'un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d'une infraction générique d'atteinte volontaire à l'environnement, appelée de leurs voeux par nombre d'interlocuteurs, dont la Conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration. » La réponse apportée par le projet de loi est décevante et s'avérera finalement peu opérationnelle pour réprimer des atteintes pourtant volontaires à l'environnement. La double condition d'intentionnalité a été critiquée par le Conseil d'État à juste titre. Au moment de commettre l'infraction, l'auteur devra savoir que son comportement entraînera une pollution, mais aussi être conscient du caractère grave et durable du dommage. Comme nous l'avons déjà évoqué, le caractère durable du dommage est très contestable, car il est très réducteur de la réalité des atteintes à l'environnement. De surcroît,

une dégradation substantielle de l'environnement, en distinguant, à l'instar de l'article 68 du projet de loi tel qu'il est issu des travaux de la commission, les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles et en retenant le même quantum des peines. Il nous faut de l'ambition dans ce domaine pour rompre avec le caractère lucratif actuel des délits et crimes environnementaux.

eau, air et sols -, en créant deux grandes infractions, l'une non intentionnelle et l'autre intentionnelle, cette dernière étant soumise à des peines plus sévères. L'équilibre ainsi trouvé permet une meilleure lisibilité du droit et répond aux critiques du Conseil d'État, qui pointait un risque d'inconstitutionnalité. L'amendement n° 370 vise à ne pas retenir la notion d'effets nuisibles graves et durables, qui permet de sanctionner la commission des infractions les plus graves. Il ne me paraît pas souhaitable, dans un premier temps et en l'absence d'étude d'impact, d'ouvrir trop largement le champ des infractions d'être concernées par ce dispositif, étant donné notamment la sévérité des peines prévues par ces nouvelles infractions, qui peuvent atteindre sept ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende. L'avis est donc défavorable. L'amendement n° 1343 rectifié L'amendement n° 1343 rectifié tend à codifier les atteintes volontaires à l'environnement dans le code pénal, plutôt que dans le code de l'environnement, ce qui est sans incidence sur la portée de ces dispositifs. En outre, les infractions proposées sont plus généralistes et n'excluent pas, notamment, les émissions dans l'air et les opérations de rejet autorisées par l'autorité administrative,

nonobstant la délivrance d'une autorisation administrative ou d'une décision administrative, lorsque celle-ci est manifestement illégale. Or cette notion d'autorisation manifestement illégale est excessivement imprécise et ne peut constituer le support d'une infraction pénale ; elle ne permet pas de circonscrire avec précision le comportement incriminé et apparaît en

Or le code de l'environnement ne contient pas de définition de cette notion ; il s'agit d'une notion scientifique qui désigne à la fois une étendue terrestre ou marine, la biodiversité qui y réside et l'environnement physique qui lui est associé, ainsi que leurs interactions. Un écosystème n'est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. La notion d'écosystème ne peut pas constituer le support d'une incrimination pénale, dès lors qu'elle est susceptible de s'appliquer à des espaces très réduits.

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir l'article 68 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. L'article 68 renforce significativement la protection judiciaire de l'environnement, à laquelle le Gouvernement est extrêmement attaché. Tout d'abord, il renforce la répression des infractions applicables en matière d'activité réglementée, lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves et durables à l'environnement. Les peines sont alors portées à cinq ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Ensuite, cet article crée un nouveau titre au sein du code de l'environnement dédié aux atteintes générales aux milieux physiques afin d'appréhender les atteintes graves à l'environnement dans leur globalité. Dans les cas les plus sévères d'atteinte intentionnelle grave et durable à l'environnement, les faits seront ainsi réprimés d'une peine de dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende, au lieu de cinq ans de prison et 300 000 euros d'amende en l'état actuel du droit. Ces évolutions permettront de réprimer à leur juste hauteur les atteintes à l'environnement les plus graves. Monsieur le président,

applicables en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Or la violation manifestement délibérée est un concept créé par la loi dite Fauchon pour protéger les personnes physiques, lorsqu'elles sont auteurs de faits dénués de causalité directe avec l'élément matériel d'une infraction volontaire. Il est important, pour ne pas mettre à bas l'édifice jurisprudentiel qui s'est construit depuis cette loi, que ce concept ne soit pas étendu à la violation « en connaissance de cause », qui est l'expression adéquate pour désigner le comportement visé par l'article L. 231-1 du code de l'environnement. Ce comportement correspond à une mauvaise foi de la qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes, mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu'il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises. Tel est l'objet du présent amendement.

afin de constituer l'infraction. Il n'est pas cohérent de devoir prouver que l'atteinte à l'environnement dure depuis sept ans- dix ans dans la version du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale -, alors que le délai de prescription est de six ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

les comportements qui ont mené à la catastrophe de l'. Pour Lubrizol, tout le monde est d'accord sur la gravité du dommage, mais, pour l'instant, les experts ne sont pas encore en mesure de définir sa durée. On ne pourrait donc pas sanctionner les fautes qui ont mené à cette catastrophe sur la base de cet article. La création d'un délit général d'atteinte à l'environnement était très attendue, mais, avec cet article, on ne répond pas à l'enjeu. On peut donc s'interroger fortement sur son utilité, même si l'esprit initial était bon. délit inapplicable, ce qui complexifiera encore le droit de l'environnement. En outre, comme nous l'avons déjà indiqué, la Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental : elle propose

qui pourrait rendre inopérant le dispositif prévu à cet article. En effet, l'article 68 dans sa rédaction actuelle, en cumulant les critères de gravité et de durabilité, reviendrait à exclure les atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. Le caractère subjectif de cette durabilité nous interroge donc beaucoup, car cela implique que nous disposions d'outils et de connaissances suffisants et adaptés lors de la survenance d'un aléa pour être en capacité de la mesurer. Pis, elle revient à exclure du champ d'application du texte des catastrophes écologiques qui ne s'étendent pas dans le temps, alors que certaines ont pourtant marqué l'histoire de notre pays. comme mes collègues, au naufrage de l', dont les experts ont établi que les atteintes n'avaient duré que deux ans, et pour cause : bénévoles et collectivités se sont chargés de faire le nettoyage. Or qui pourrait considérer ici que ce naufrage n'a pas eu des atteintes très graves sur l'environnement ? Si, demain, une catastrophe similaire se produisait, serait-elle donc exclue du champ d'application de cet article ? Par cet amendement, nous souhaitons retenir l'adjectif « significatifs », et non pas « durables », car c'est, selon nous, la seule condition pour rendre le dispositif opérant.

En effet, cet article, qui concerne la pollution aquatique, s'applique sans que le parquet ait à faire la preuve d'une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou d'endommager les milieux. Il convient donc, pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de souligner que cet article continue d'être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l'article 68 du présent projet de loi.

amendement vise à sécuriser le dispositif de l'article 68. Tel que résultant des travaux de commission, ce texte risque de faire peser sur les agriculteurs des risques juridiques particulièrement importants. importants. Il est donc proposé de revenir au texte de l'Assemblée nationale, tout en maintenant la simplification opérée en commission entre atteintes non intentionnelles et atteintes intentionnelles à l'environnement. Tel est l'objet de cet amendement, Pour qu'une sanction soit réellement dissuasive, elle doit être proportionnée. Par cet amendement, nous proposons donc d'établir une corrélation entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de l'amende. Concrètement, nous souhaitons que le montant maximum d'une sanction applicable à une entreprise puisse être porté à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes. En effet, pour certaines grandes multinationales, dont le chiffre d'affaires peut s'exprimer en milliards, nous ne voyons pas comment une sanction de 4,5 millions d'euros, comme le prévoit l'article 68, pourrait être dissuasive. Certes, l'article prévoit aussi que ce montant peut être porté au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction, mais cette notion nous semble pouvoir prêter à interprétation. Une entreprise pourrait très bien réussir à prouver qu'elle n'a pas tiré d'avantage direct de telle ou telle infraction. Nous pensons que laisser au juge la possibilité de fixer le montant d'une sanction en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise est la solution la plus efficace. dans notre droit de préciser la manière dont la sanction doit se calculer et ce qu'il faut retenir ou non dans la comptabilité de l'entreprise reconnue responsable de la commission d'une infraction. Encore une fois, le quantum de la peine n'est pas excessif. Je rappelle que la convention judiciaire d'intérêt public, introduite en 2016, et particulièrement efficace depuis cette date,

exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l'article L. 231-1 du code de l'environnement, créé par l'article 69 de ce projet de loi. Il s'agit donc ici d'éviter qu'une personne, en se prévalant d'une telle autorisation, puisse échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation. Là encore, je suis étonnée de l'avis défavorable de la commission, puisqu'il s'agit d'une disposition de bon sens. En effet, on ne comprendrait pas qu'une entreprise reconnue coupable d'une infraction au code de l'environnement puisse opposer une autorisation irrégulière pour se soustraire aux obligations, qui incombent à toute personne physique ou morale, de réparer le dommage causé.

l'action judiciaire par l'action administrative. Il faut rappeler qu'en présence d'une autorisation administrative illicite le juge pénal peut néanmoins condamner.

Pour nous, imposer une durée, qu'elle soit de dix ou de sept ans, rend inopérant ce texte et serait même, de l'avis de certains experts, contraire au droit européen. Nous tenons à rappeler que le fait de caractériser une durée nécessite d'avoir les outils et les connaissances nécessaires au moment de la survenance de l'atteinte. Cela nécessite également une capacité d'expertise, dont les services de la police de l'environnement, du ministère public ou les victimes ne disposent pas directement. Quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer de sept ans ou de dix ans, il sera aisé de la contredire et, ainsi, en semant le doute, d'éviter toute condamnation. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cette référence à la durabilité d'une atteinte. L'amendement

sera sans doute l'oeuvre d'une jurisprudence soutenue durant plusieurs années, à différents niveaux, y compris au niveau européen. Nous avons donc le devoir absolu d'éclairer

qu'il n'a jamais eu l'intention de commettre délibérément, mais qui a été causé par son activité ? De la même façon, nous avons besoin d'avoir plus de précisions sur l'intentionnalité. Je sais que la jurisprudence, dans bien d'autres domaines, reconnaît une intentionnalité là où, manifestement, il n'y en a pas. C'est une intentionnalité du fait de la responsabilité inhérente à l'exercice

pend au nez, si vous me permettez cette expression triviale, de tous ceux qui ont encore, dans notre pays, le courage d'entreprendre et qui risquent, par ce titre VI, d'en être fortement dissuadés.

Est occulte l'infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte. En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription, dans la mesure où les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d'infraction occulte ou dissimulée. En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra, de toute façon, pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. Les deux

l'amendement n° 1481. Au vu de l'urgence environnementale et climatique à laquelle nous devons faire face, nous considérons qu'il n'est plus possible aujourd'hui de négocier avec la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons renforcer notre arsenal juridique pour sanctionner les conduites à risque les atteintes à l'environnement. Nous estimons que l'inscription d'un délai de prescription de douze ans dans la loi n'est pas du tout conforme à cet esprit. D'un côté, le texte prévoit qu'une atteinte durable ne sera considérée comme telle que si elle dure plus ou de dix ans. De l'autre, on nous impose un délai de prescription de douze ans. Nous avons le sentiment que tout est mis en oeuvre pour que le dispositif retenu soit le moins contraignant et applicable possible. Par cet amendement, nous demandons donc la suppression de ce délai de prescription tel qu'il a été introduit par la commission.

Il vise à renforcer les sanctions applicables aux faits prévus à l'alinéa 21 lorsque les infractions sont commises par une entreprise. Nous estimons en effet indispensable d'établir une corrélation entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de l'amende qui lui sera appliquée, et ce afin de rendre les sanctions réellement dissuasives.

qu'il est préférable de réserver aux crimes susceptibles d'être jugés par des juridictions pénales internationales. La rédaction proposée est source de complexité, car elle distingue les milieux et ne retient pas une ligne de partage claire et univoque entre les infractions non intentionnelles et celles commises de façon intentionnelle.

l'amendement n° 907 rectifié. Ses auteurs proposent de ne pas retenir le délit générique de pollution des sols adopté par la commission, mais de le rattacher aux prescriptions administratives relatives à la gestion et à la prévention des déchets. Cette formulation permet d'extraire les activités agricoles du champ des infractions portant des atteintes graves et durables à la qualité des sols. S'il convient, comme le soulignent les auteurs de cet amendement, de protéger les agriculteurs de tout risque d'incrimination

Abandon du projet EuropaCity, abandon de la construction du terminal 4 de Roissy, assignation d'ArcelorMittal, recours contre le chlordécone ou encore combat contre la chasse à la glu : les exemples ne manquent pas pour illustrer le dynamisme et la pugnacité des associations de défense de l'environnement et de toutes celles et de tous ceux Contre-pouvoirs salutaires pour les uns, empêcheurs de tourner en rond pour d'autres, les associations jouissent dans notre pays d'une place et d'un rôle reconnus, qui font d'elles des composantes essentielles de notre démocratie. Les associations de protection de l'environnement ont fait preuve de leur engagement. L'agrément leur permet d'agir en justice devant les tribunaux administratifs, de se constituer parties civiles pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires. Nous souhaitons, au vu de l'évolution des pratiques constatées, étendre leurs prérogatives. Comme le souligne très justement France Nature Environnement, cet élargissement est d'autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd'hui obstacle à une action des associations devant le juge civil, puisque l'amende administrative remplace l'amende pénale.

à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Nous sommes d'accord sur la finalité.

ils visent à permettre aux associations non agréées déclarées depuis au moins cinq ans d'engager cette action civile. Je comprends l'objectif visé par ces amendements, qui est de sécuriser le droit à agir de ces associations en matière civile. J'observe toutefois que l'adoption de ces amendements n'aurait pas que des avantages. La jurisprudence reconnaît déjà la recevabilité des actions des associations devant les juridictions civiles pour la défense d'intérêts collectifs, dès lors que ces intérêts entrent dans leur objet social. Ces associations peuvent agir, qu'elles soient agréées ou simplement déclarées, même depuis moins de cinq ans, et indépendamment de toute infraction pénale. Il suffit qu'elles justifient d'un intérêt à agir au nom d'un intérêt collectif, lequel est déterminé par leur objet social. l'extension de l'habilitation législative sollicitée n'apparaît pas nécessaire. Elle pourrait même être contre-productive, car il y a un risque qu'elle soit interprétée comme une limitation du pouvoir d'action de ces associations. Je m'explique : la définition de l'habilitation à agir est plus limitée que celle qui résulte de la jurisprudence ; par ailleurs, pour les associations non agréées, l'amendement subordonne leur action à la condition d'être déclarées depuis cinq ans au moins, alors que la jurisprudence ne l'impose pas. J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

et à ceux-ci de pouvoir la recueillir. C'est une mesure de simplification, tant pour le bureau d'ordre du parquet que pour les victimes, puisque les plaintes seront regroupées dans une seule procédure. Les victimes identifiées, souvent oubliées à l'issue de l'enquête, pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives ou aux poursuites pour demander réparation. Il s'agit d'améliorer l'accès à la justice pénale en la simplifiant, en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile. il vise à autoriser les inspecteurs de l'environnement, les autres fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre de police spéciale du code de l'environnement

Quel est l'avis du Gouvernement ? En fait, il s'agit déjà du droit existant. En effet, les inspecteurs de l'environnement peuvent déjà recueillir des plaintes ou déclarations des victimes des infractions prévues par le code de l'environnement, en application de l'article L. 172-8

des marchés publics les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour des atteintes à l'environnement. Certes, les décisions que nous avons prises aujourd'hui et le rejet d'un certain nombre d'amendements font que, finalement, cette loi apparaît très tiède créer un certain nombre de nouvelles infractions d'atteinte à l'environnement. Néanmoins, afin d'appuyer cette toute petite avancée, il est primordial que les personnes responsables de tels agissements et qui ont été condamnées définitivement ne puissent pas accéder aux marchés publics. Comparaison n'est certes pas raison, mais, par exemple, le récent gifleur du Président de la République a été interdit d'exercer toute fonction publique pour dix années. N'y a-t-il pas une forme de logique dans le fait de ne pas vouloir contracter avec des personnes qui sont coupables de crime ou de délit de mise en danger de l'environnement, au même titre qu'un homme qui trouble l'ordre public ? La question sous-tendue par ces amendements est simple : souhaitons-nous céder des activités relatives aux marchés publics à des personnes ayant été condamnées pour atteinte grave à l'environnement ?

Mme la ministre.

et les sanctions à visée dissuasive. Le présent amendement a donc pour objet de permettre au juge de condamner les personnes morales responsables d'écocide aux peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du code pénal, telles que l'interdiction d'accès aux marchés publics. Il a également pour objet de créer deux circonstances aggravantes. Ainsi, l'atteinte à la santé des personnes, comme c'est le cas avec le chlordécone, constituerait, si cet amendement si cet amendement était adopté, un facteur aggravant de l'infraction. Cela permettrait de décorréler l'atteinte à l'environnement de l'atteinte aux populations humaines, sans pour autant exclure les sanctions prévues. Par ailleurs, cet amendement vise à ce que le caractère irréversible de l'atteinte à l'environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles que les infractions préexistantes au code de l'environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations dans lesquelles la réparation ou la remise en état sont rendues impossibles par l'ampleur de l'atteinte. Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l'environnement, en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d'ores et déjà

Ce franchissement peut nous conduire vers un point de basculement caractérisé par un processus d'extinction irréversible d'espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques nocives pour l'humanité. Le dernier rapport sur l'état de l'environnement en France énonce « qu'outre le fait de constituer un cadre d'analyse novateur, l'approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d'actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et citoyennes, ainsi qu'aux décideurs et décideuses, une compréhension plus globale de la situation nationale ». L'introduction des limites planétaires dans le droit français vise à protéger l'équilibre des milieux naturels et l'habitabilité des territoires, une manière novatrice de concevoir le droit environnemental afin d'offrir

au titre du développement durable a pour ambition d'inscrire ces nouvelles références au coeur de la politique environnementale française, comme le recommandent les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Quel

Cette notion, qui ne fait pas encore l'objet d'un consensus parmi la communauté scientifique, pose plusieurs problèmes, notamment la fixation de seuils qui détermineraient les limites à ne pas dépasser. Il n'est pas opportun d'élever la protection des limites planétaires au titre des engagements à satisfaire par la France au titre du développement durable, dans la mesure où cette notion

est ici question de compléter l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans lequel figurent, parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable, de grands principes, tels que le principe de précaution, le principe de prévenir et de corriger les atteintes, le principe pollueur-payeur, ou encore le principe de participation du public et le principe de non-régression.

Cet amendement fait suite à notre précédent amendement visant à introduire la notion de limites planétaires dans notre droit. Il tend à inscrire la définition des limites planétaires dans notre législation afin de garantir le respect de l'équilibre des milieux naturels et le développement durable et juste de l'humanité, conformément au mandat de la Convention citoyenne pour le climat. Cette définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, les apports en azote et phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d'usage des sols, l'acidification des océans, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'usage de l'eau douce, la dispersion d'aérosols atmosphériques, la pollution chimique imputable aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l'équilibre des milieux naturels, ainsi qu'avec le développement durable et juste de l'humanité. Je tiens à rappeler, en ce sens, que la France dépasse déjà actuellement six des neuf limites planétaires. Cet amendement est donc une invitation à faire un état des lieux de notre action en matière environnementale, ainsi qu'à remettre en question nos modes de consommation et de production. La commission

Esther Benbassa. La procédure du référé-liberté, telle que définie à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permet une intervention du juge administratif des référés en moins de quarante-huit heures, sous les deux conditions que nous connaissons la demande doit présenter un caractère urgent et elle doit démontrer que l'intervention du juge est nécessaire « à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Ce type de référé s'applique notamment au droit d'asile, au droit de propriété, au droit de grève, au droit syndical, ou encore au droit de mener une vie familiale normale, ces droits entrant tous dans la définition classique des libertés fondamentales. La question de l'extension du référé-liberté visant à intervenir en urgence pour la prévention d'atteintes à l'environnement n'est pas nouvelle. Ainsi, la mission flash d'information menée par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier a permis des avancées concernant le contentieux de l'environnement.

consacrés par la Charte de l'environnement de 2004 dans le champ d'application du référé-liberté. L'importance de la protection de l'environnement justifie un tel amendement. Son adoption assurerait la possibilité de protéger l'environnement dans des situations d'extrême urgence.

je l'ai dit précédemment, la volonté du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est de renforcer autant les moyens du juge en matière de protection de l'environnement que l'arsenal pénal et les sanctions

La sanction de la récidive est ancrée dans notre droit pénal à bien des égards. Nous pouvons classiquement citer le cas de l'infraction de vol, assimilée à celle d'escroquerie ou d'abus de confiance au regard de la récidive.

une proposition du rapport de la mission d'information flash, présentée lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Il vise à assimiler différentes infractions au regard de la récidive, afin de mieux réprimer les comportements récidivistes en matière environnementale et, ainsi, de renforcer l'effet dissuasif des sanctions proposées. Ce mécanisme existe d'ores et déjà en droit pénal français. Ce n'est donc pas un non-sens de l'envisager pour la protection de l'environnement.

Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a posé une première pierre dans l'extraterritorialité de la réglementation environnementale, afin de lutter contre la délocalisation des pollutions à l'aide de dispositifs juridiques permettant de sanctionner les entreprises qui profitent de législations moins contraignantes pour commettre à l'étranger des infractions répréhensibles en France. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite adapter les dispositions applicables en matière de corruption à la matière environnementale. Son objectif est de faciliter la poursuite des délits environnementaux commis par des sociétés françaises à l'étranger, en simplifiant les conditions d'engagement des poursuites de ces délits par le juge français suivre l'exemple des infractions de corruption pour la procédure- requête du ministère public, double incrimination, plainte de la victime ou dénonciation de l'État d'étendre l'extraterritorialité aux filiales étrangères des sociétés mères françaises qui commettraient des infractions de façon intentionnelle. Afin d'améliorer la responsabilité civile des entreprises pour leurs activités à l'étranger, le présent amendement vise à mettre à la charge de certaines sociétés une obligation de vigilance environnementale, sur le modèle de l'obligation de vigilance anti-corruption de la loi Sapin II.

elle nous appartient à tous. Il convient de lutter ardemment contre la pollution de nos entreprises, sur notre territoire et à l'étranger. Je

En 2011, un rapport parlementaire fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a mis en lumière, au niveau national, les conséquences économiques, sanitaires et environnementales de l'utilisation du chlordécone- pesticide organochloré -entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique, pour lutter contre le charançon du bananier. Alors que, dès 1966, les dangers pour la santé humaine et animale de ce pesticide étaient connus, son utilisation s'est poursuivie jusqu'en septembre 1993, sur le fondement de deux dérogations successives accordées par le ministère de l'agriculture, à la demande des professionnels du secteur. Il s'agissait là d'un choix politique et de société, un choix productiviste et économique d'autoriser le chlordécone afin d'être encore encore et toujours plus compétitif. Ce productivisme à outrance est la cause de nombreuses conséquences néfastes pour l'environnement et pour l'homme : pollution des sols, taux élevé des cancers de la prostate, notamment. Face à ce que l'actuel Président de la République appelait en 2018 un « scandale environnemental il revient maintenant au Gouvernement, après les travaux menés par le Parlement, de se pencher sérieusement sur l'urgente question de l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises, pour une appréciation des responsabilités publiques comme privées. Il s'agit aujourd'hui de sanctionner

? Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur l'impact sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique. Ses auteurs souhaitent que ce rapport permette de faire le point sur les responsabilités, publiques comme privées, dans la prolongation de son autorisation. Je ne crois pas qu'un rapport au Parlement soit le meilleur vecteur d'information

très abondante, notamment sur le plan scientifique. S'agissant de la question de la responsabilité, elle a été examinée en profondeur par le rapport de la commission d'enquête parlementaire

Dans les ICPE ou les ouvrages hydrauliques, le recours aux drones rend plus opérationnelle et efficace la constatation d'écarts à la réglementation ou de dommages à l'environnement. Ainsi, l'utilisation de drones permettra de faciliter la constatation des pollutions dans les milieux naturels, des emprises et volumes de stockage de produits dangereux ou de déchets, et des dépôts de déchets volontairement dissimulés. Cet amendement vise à apporter des garanties utiles en matière de protection de la vie privée et de gestion des enregistrements, afin de donner un cadre rigoureux rigoureux à l'utilisation de ces drones. Il est prévu de limiter l'usage des drones au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement et des ouvrages hydrauliques. Cette restriction permet de s'écarter des domiciles et lieux de promenade usuels des particuliers et, ainsi, de donner plus de garanties sur l'absence de collecte de données personnelles. également prévu de limiter le recours aux drones aux seuls cas des contrôles administratifs, en respectant une information préalable de l'exploitant ; de limiter l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées à cette fin ; de restreindre l'usage des drones au recueil d'informations qui serait manifestement plus et plus long lors du contrôle au sol. En ce sens, l'amendement s'inscrit dans l'esprit des adaptations établies en commission en prévoyant des conditions plus précises. le rapporteur. Ce sous-amendement vise à conserver le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images, ainsi que de données physiques ou chimiques, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission par des amendements communs avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette autorisation serait délivrée par décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente, qui déterminerait son périmètre et sa période de validité, qui ne pourrait excéder un mois, ainsi que ses finalités.

Cet amendement vise à habiliter les agents chargés de la police des pêches maritimes à employer des drones dans le cadre de l'exercice de leur mission de police administrative. Plusieurs expérimentations de surveillance des pêches maritimes par drones sont menées actuellement par les forces de la fonction garde-côtes. Elles démontrent l'efficacité de ces technologies pour rechercher et constater les infractions au code rural et de la pêche maritime. Les drones ont une complémentarité indéniable avec les moyens nautiques déjà employés par les unités de contrôle et ils peuvent couvrir des distances importantes en un temps limité. Il est nécessaire de clarifier la possibilité pour les agents chargés de la police des pêches maritimes de recourir à ces technologies dans le cadre de leurs contrôles administratifs, en complément des moyens traditionnels de surveillance et de contrôle en mer. Cet usage sera limité aux polices en mer ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de la juridiction française. Les usages pour les contrôles terrestres sont exclus. Les délais d'effacement des données sont encadrés. Enfin, les atteintes à la liberté des personnes sont prévenues, notamment par l'interdiction de la visualisation d'images de locaux affectés à des usages privés ou d'habitation, en prévoyant l'information préalable du public susceptible d'être survolé.

une proposition sur le référé spécial environnemental introduite par une mission d'information flash sur ce sujet. Cet article visait à élargir le champ d'application du référé pénal spécial, prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement, à l'ensemble des dispositions prévues dans le code de l'environnement et le code forestier, l'ensemble des délits à caractère environnemental qui entrent dans le champ de compétence des nouveaux pôles juridictionnels environnementaux, institués par l'article 15 de la loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Notre groupe estime que la suppression de cette disposition par la commission sénatoriale est regrettable. Nous en proposons donc Cet amendement vise à rétablir un article supprimé par la commission. Les juges des libertés et de la détention ne se saisissent que très rarement de cette procédure éloignée de leur coeur de métier. Les acteurs de la protection de l'environnement n'empruntent pas

Aujourd'hui, la récidive est punie de 3 000 euros, ce qui paraît suffisamment dissuasif pour une amende qui frappe principalement les ménages. Pour cette raison, l'avis est défavorable.

cet amendement avec le Gouvernement. Je tiens à remercier les services du ministère de la transition écologique, en particulier la direction générale de la prévention des risques, pour cette collaboration. Cet amendement vise à réécrire l'ensemble de l'article 71 pour préciser les missions et compétences des agents du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques.

La commission d'enquête du Sénat, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Nicole Bonnefoy et Christine Bonfanti-Dossat, avait souhaité la création de ce bureau d'enquêtes plutôt que celle d'une autorité indépendante.

les deux chambres du Parlement. Dans le détail, cet amendement tend à insérer un titre préliminaire au sein du livre V du code de l'environnement : la section 1 définit la procédure et les missions de ce bureau la section 2 définit les pouvoirs d'investigation du bureau et l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire, ainsi que les conditions d'indépendance de ce bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ; la section 3 définit les conditions d'exercice du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire

parole est à Mme la ministre. Cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures prévues par le code général des impôts avec celles du code de l'environnement pour protéger les riverains des sites Seveso seuil haut face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels. Les PPRT peuvent prescrire des travaux de renforcement des logements pour protéger les occupants des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut. Ce sont ainsi près de 16 000 logements qui doivent faire l'objet de travaux de renforcement. L'accompagnement de l'État se matérialise un crédit d'impôt aux contribuables propriétaires des logements de 40 % des dépenses éligibles tel que prévu par le code général des impôts. Le code de l'environnement prévoit une participation des exploitants industriels à l'origine du risque et des collectivités territoriales à hauteur de 50 % des travaux nécessaires. Toutefois, ledit code réserve ce financement aux « personnes physiques propriétaires de logements », excluant donc les autres contribuables, notamment les sociétés civiles immobilières gérant, par exemple, des HLM.

unique pour certains délits en matière d'environnement et d'urbanisme en procédant à trois modifications : premièrement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre I du livre IV du code de l'environnement ; deuxièmement, en étendant la compétence du juge unique à l'ensemble des délits prévus par le code de l'urbanisme, alors qu'elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts » ; troisièmement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime. Il s'agit d'adaptations

Un rapport du Conseil général de l'économie de janvier 2020 est venu dresser un bilan mitigé de l'application de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des entreprises. Il a notamment pointé la nécessité de mieux définir son champ d'application, aujourd'hui si imprécis que l'administration n'est même pas en mesure de déterminer les entreprises qui y sont réellement assujetties.

Nous considérons que l'application efficace du devoir de vigilance constituera un avantage compétitif pour les entreprises françaises vis-à-vis de leurs homologues européennes, dans la perspective d'une potentielle reprise des principes de la loi française à l'échelle européenne. C'est la raison pour laquelle nous avons repris à notre compte la proposition formulée par le Conseil général de l'économie. Nous ne souhaitons pas revenir sur cet équilibre, qui concilie l'amélioration de la portée du droit de l'environnement et le renforcement de la sécurité juridique. La commission est donc défavorable

du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport doit notamment présenter l'incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l'environnement et constatées par les agents habilités à cet effet sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l'environnement. L'évaluation des politiques publiques est tout de même l'une des prérogatives du Parlement. En ce sens, cette disposition est une bonne chose. Nous regrettons une fois de plus que la commission sénatoriale

ministre. Cet amendement vise à rétablir l'article 76 de l'Assemblée nationale, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l'environnement prévues dans les différents codes et textes non codifiés. Il est utile de se demander si une évolution de notre codification est nécessaire au regard de l'accroissement des dispositions en lien avec la protection de l'environnement. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite donc le rétablissement

Sur le fond, on perçoit mal l'avantage qu'il y aurait, du point de vue de la lisibilité du droit, à regrouper dans un code unique des dispositions pénales qui tirent les conséquences de la violation de règles posées dans de multiples codes, d'autant que, si le Gouvernement l'estime nécessaire, il lui est loisible de déposer un projet de loi à cette fin, l'exposé des motifs et l'étude d'impact permettant

Le cabinet I4CE considère que « le principal problème vient du mode de construction et du manque de pilotage de la stratégie. La SNBC est un document technocratique, pas politique.

Une bonne coordination entre ces organismes permettrait d'assurer un meilleur suivi des mesures prises et des corrections à apporter en termes de budgets carbone, par exemple, pour respecter la trajectoire fixée par la SNBC. Il est aussi nécessaire d'assurer la cohérence entre le pilotage national et les initiatives décentralisées des acteurs dans les territoires. Un dialogue entre les différentes parties prenantes est donc nécessaire pour réussir la transition écologique, laquelle suppose la reconversion de nombreux secteurs d'activités. Enfin, et le mouvement des « gilets jaunes » qui avait conduit au gel de la trajectoire de la contribution carbone en 2019 est là pour nous le rappeler, sans évaluation des impacts sociaux des mesures en termes de pouvoir d'achat, de déplacements ou d'emplois, la transition écologique est condamnée à échouer, faute d'acceptabilité sociale. sociale. Cet amendement vise précisément à répondre à la défaillance du pilotage de la SNBC en demandant au Gouvernement un rapport sur son contenu et sur la possibilité de confier son organisation au haut-commissariat au plan- dont on se demande à quoi il sert -ou à tout autre organisme compétent.

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir l'article 76 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui avait fait l'objet d'un large accord transpartisan. Cet amendement vise ainsi à confier à la Cour des comptes la mission d'évaluer annuellement la mise en oeuvre du présent texte. Nous partageons tous l'enjeu et l'intérêt l'enjeu et l'intérêt de veiller en toute transparence à la mise en oeuvre rapide des mesures prévues dans ce projet de loi. Cette mission d'évaluation relève bien du champ de compétence de la Cour des comptes au titre de l'article 47-2 de la Constitution. En outre,

par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la SNBC à annexer au projet de loi de programmation énergie et climat. Cette première loi de programmation, à adopter avant le 1 juillet 2023, 2023, fixera les grands objectifs et les priorités d'action de la politique climatique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Ce rapport-bilan viendra en complément de l'étude d'impact du projet de loi. Il vise à donner au Parlement

des lames de fond les plus majeures qui va impacter notre pays au cours du siècle à venir. n° 2182, je rappelle que la commission a adopté un amendement visant à confier au Haut Conseil pour le climat la mission d'évaluer la mise en oeuvre du projet de loi. Je rappelle également que le Président de la République a fait le choix, après la crise des « gilets jaunes d'investir le HCC d'un rôle spécifique d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Nous estimons qu'il revient au HCC la responsabilité d'évaluer une loi devant permettre à la France de respecter l'accord de Paris de 2015. En tout état de cause, le manque de moyens du Haut Conseil ne saurait justifier le recours, à titre principal, à l'expertise de la Cour des comptes. Lors du dernier projet de loi de finances, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait d'ailleurs proposé un amendement tendant à augmenter substantiellement les moyens humains du HCC. Nous n'avons pas été écoutés par le Gouvernement, madame la ministre : à lui d'assumer ses choix ! C'est bien le Président de la République qui a souhaité faire du HCC une instance d'expertise climatique. Par ailleurs, avec la commission des affaires économiques, nous avons souhaité supprimer le deuxième alinéa de l'article 76, qui prévoyait un rapport annexé à la « loi quinquennale » énergétique prévue à compter de 2023. Nous avons considéré que ce rapport était superfétatoire, puisque cette loi doit déjà faire l'objet,

des négociations sur la répartition de l'effort entre les secteurs et les différents États membres. Bien évidemment, la France se mobilisera pour faire sa pleine et juste part de cet effort. Il serait anticipé de quantifier cet objectif dès aujourd'hui dans la loi.

? Vous souhaitez que le Haut Conseil pour le climat remette un rapport évaluant l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Votre demande me semble déjà satisfaite. En application de l'article 68 de la loi Énergie-climat, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport concernant la contribution des PCAET et des Sraddet aux politiques de transition écologique et énergétique- il sera remis au Parlement d'ici à la fin de l'année.

des collectivités territoriales créé au sein du CNTE, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en oeuvre la stratégie nationale bas-carbone. Il s'inscrit dans l'esprit des travaux réalisés dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, qui a proposé de renforcer de centraliser l'évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale et qui a souligné la nécessité de disposer d'un organisme indépendant à l'égard de l'État. Cet observatoire permettra d'opérationnaliser la SNBC, en impliquant tous les acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique en créant un cadre légal unifié. Il rendra ainsi beaucoup plus visible la part prise par les collectivités dans la transition écologique pour la valoriser.

multipartites, en impliquant pleinement les secteurs les plus émetteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au travers de ce mécanisme de feuilles de route sectorielles, les députés avaient fait le choix de la responsabilisation de toutes les parties prenantes, en créant un cap de négociation, dans laquelle les divers acteurs concernés pouvaient prendre des engagements pour atteindre collectivement l'objectif de baisses d'émissions du secteur. Il s'agit bien là de travailler sur la synergie entre les actions des uns et des autres, afin de surmonter les éventuels freins et blocages qui limiteraient l'atteinte de nos objectifs climatiques communs. Le fait que le Sénat ait souhaité supprimer cette disposition, qui visait à une plus grande flexibilité et adaptation de la mise en oeuvre de la SNBC m'interroge, puisque c'est exactement ce que les acteurs demandent, à savoir plus de flexibilité et de synergies. La rédaction de cet amendement n'est pas parfaitement identique à ce qui a été voté

comme les comités stratégiques de filières. Elle s'appliquera en revanche aux secteurs les plus émetteurs n'ayant pas encore adopté de feuille de route climatique. Avec la commission des affaires économiques, saisie pour avis, nous avons considéré que le pouvoir exécutif n'avait nullement besoin du mandat du Parlement pour engager des échanges avec les parties prenantes des filières économiques et les représentants des collectivités territoriales, qui plus est dans la perspective de mettre au point des feuilles de route, dispositif par nature non normatif.

de produits contenant des micropolluants, y compris les produits du quotidien. Ces produits sont nocifs pour l'environnement et la santé. Ils font l'objet de listes de vigilance en France et au sein de l'Union européenne. Ce rapport permettrait d'appliquer enfin le principe « pollueur-payeur et d'examiner la pertinence d'un éventuel élargissement de la redevance pour pollutions diffuses perçue par les agences de l'eau. Ces nouvelles ressources pourraient financer la lutte contre les micropolluants. Une telle redevance pourrait en outre inciter les industriels à une écoconception de leurs produits.

ils donnent lieu à des phénomènes de bioaccumulation, c'est-à-dire des accumulations dans les tissus de l'organisme. Actuellement, en Europe, 110 000 substances chimiques circulent dans notre environnement.

dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation. Il est également prévu que l'application du texte fasse l'objet d'une évaluation par l'Opecst. Si nous avons souhaité confier au HCC la responsabilité d'évaluer l'application de la loi, rien n'empêche pour autant que des structures parlementaires se saisissent parallèlement de cette tâche. Faut-il pour

dont les missions seraient d'évaluer et d'assurer le suivi des incidents et accidents, d'émettre des préconisations à toute entreprise faisant usage de produits chimiques, y compris dans le domaine agroalimentaire ou l'agriculture. Nous avons tous en mémoire les accidents liés au stockage de produits chimiques et même au fonctionnement de certaines entreprises, comme AZF en 2001,

de la commission ? Cet amendement vise à introduire une énième demande de rapport au sein de ce projet de loi. Nous disposons d'autres moyens pour évaluer l'opportunité de créer cette autorité de sûreté chimique. Par ailleurs, d'autres établissements publics et autorités interviennent déjà sur ce sujet.

Madame la ministre, du volet agricole de la feuille de route économie circulaire. En février 2020 a ainsi été intégrée au Géoportail de l'IGN une nouvelle carte, qui donne la description des différents types de sols. Le travail se poursuit, pour être encore plus précis,

Au cours de l'agenda 2030, dix-sept objectifs de développement durable, les ODD, ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement durable dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation. À l'instar des études d'impact devenues obligatoires pour chaque projet de loi examiné par le Parlement, il est aujourd'hui indispensable de rendre obligatoire une partie consacrée aux ODD que la France s'est engagée à atteindre d'ici à 2030. Cette partie aurait pour fonction de reprendre une à une les dispositions du projet de loi et d'indiquer, pour chacune d'entre elles, l'ODD ou les ODD auxquels elle est censée répondre. Cela serait très positif et nous permettrait d'avoir une lisibilité toute simple sur chaque projet de loi. À chaque article, il serait indiqué à quel ODD il répond. l'avis de la commission ? Les objectifs de développement durable doivent effectivement constituer une boussole dans la conduite de nos politiques publiques. Il est certain nous devons nous appuyer plus largement sur cet outil, notamment dans l'élaboration des politiques publiques. Faut-il pour autant intégrer dans tout projet de loi une partie consacrée à l'évaluation des dispositions dudit projet au regard des objectifs de développement durable ?

du Gouvernement ? Votre assemblée a approuvé le 17 mai dernier le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son article 2 prévoit qu'avant le 1 juin de chaque année le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur la cohérence des politiques publiques françaises avec les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations unies. Ces dispositions apportent une réponse à l'évaluation des politiques publiques au regard des ODD. Considérant que votre amendement

Dans ces pays, un groupe de scientifiques appartenant à toutes les disciplines est mobilisable dès la survenue d'un accident ou au commencement d'une crise. Cet organe est chapeauté par un scientifique en chef- je pense à cet égard au scientifique en chef du Québec, que nous avons auditionné à l'Opecst -capable de mobiliser tous les chercheurs dont il a besoin pour documenter la crise en question et conseiller le Gouvernement. Plutôt que d'envisager la mise en place d'un conseil scientifique uniquement en cas de crise grave et, donc, avec un délai de réponse, il serait plus pertinent de prévoir ce type d'instance pérenne et susceptible de se rendre disponible immédiatement.

Il ne me semble pas opportun de multiplier les instances d'expertise sur le climat. Le morcellement des moyens contribue souvent à l'affaiblissement des structures. Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

l'exemple de la crise sanitaire le démontre, l'exécutif est en mesure de réunir très rapidement un conseil scientifique pour éclairer ses décisions. Je ne vois pas l'urgence qui obligerait à mettre en place ce que vous souhaitez. Par ailleurs, je tiens à le souligner, pour ce qui concerne le climat, le Haut Conseil pour le climat a pour mission de conseiller les décideurs politiques sur les orientations de moyen et long terme, d'évaluer l'action climatique française et de recommander, le cas échéant, des actions correctrices. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Cette partie du projet de loi touche directement au coeur de l'une des compétences des élus locaux : la capacité de définir leur propre projet de territoire. Cette compétence me tient particulièrement à coeur, alors que nous débutons en parallèle l'examen du projet de loi 4D, qui promet justement la décentralisation et la différenciation. La proposition que nous fait le Gouvernement dans ce chapitre est la suivante : un double objectif de réduction de l'artificialisation des sols avec, d'une part, une réduction de moitié du rythme d'artificialisation en dix ans et, de l'autre, une cible de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. Le coeur du dispositif rend obligatoire l'intégration de ces objectifs dans les documents de planification des collectivités. Pour résumer cette mécanique complexe, les Sraddet devront inscrire cet objectif de réduction d'au moins 50 % du rythme d'artificialisation, ainsi qu'une une répartition entre les différentes parties du territoire régional. La région fixera donc aux collectivités de niveau inférieur des objectifs chiffrés de réduction, charge ensuite aux SCoT et aux PLU de les traduire. La commission a jugé, et j'en suis moi-même convaincu, que cette approche centralisée, uniforme et prescriptive n'était pas la bonne. Pour autant, comprenez bien, madame la ministre, que nous partageons votre ambition de lutter contre l'étalement urbain et la dégradation des sols. Les collectivités sont d'ailleurs déjà fortement engagées, la plupart du temps, dans cet effort, et les outils sont en partie déjà là. Avant-hier, en séance publique, sur le chapitre consacré aux transports, la ministre Emmanuelle Wargon disait : « La condition de l'acceptabilité des décisions, c'est la différenciation territoriale. C'est cette acceptabilité, cette différenciation que notre commission a tenté d'insuffler aux chapitres relatifs à l'artificialisation des sols. Nous avons d'abord replacé le Sraddet dans son rôle d'orientation générale. Nous ne souhaitons pas en faire un grand répartiteur des droits à construire, au mépris de la compétence des communes et des EPCI en matière d'urbanisme. Nous avons donc souhaité que les SCoT et les PLU puissent avoir une plus grande marge de manoeuvre dans la manière dont ils déclinent l'orientation régionale. Nous avons ensuite renforcé la territorialisation au niveau infrarégional en encadrant les critères qui permettront aux collectivités de justifier leurs propres objectifs les enjeux propres à la ruralité, les besoins économiques, les trajectoires passées, les projets au service de tout un territoire. En parallèle et en contrepartie de cette plus grande flexibilité, nous avons souhaité montrer que les collectivités agissaient en responsabilité, en renforçant la logique de bilan et d'évaluation des documents d'urbanisme. Je pense que nous pouvons tous, des travées, nous retrouver dans ces objectifs de territorialisation et de différenciation sans qu'ils mettent aucunement en péril, madame la ministre, l'ambition que nous partageons. La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Je tiens à remercier, avant de commencer ce chapitre, les sénateurs et sénatrices d'avoir choisi d'aller dans le sens de la réduction du rythme d'artificialisation

faire de façon opérationnelle. Vous le savez, l'artificialisation des sols est un fléau, dont nous payons le prix très régulièrement. Malheureusement, les dernières inondations que nous avons connues sur notre territoire montrent le travail qui reste à Je sais l'attachement des collectivités et des exécutifs locaux que vous représentez à leur pouvoir décisionnaire en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. J'y suis également très attachée, comme le Gouvernement. Gouvernement. Nous ne cherchons pas dans cette loi à imposer une forme de centralisme en matière d'aménagement du territoire. Au contraire, nous confions aux différents échelons territoriaux la mission de mettre en oeuvre et d'atteindre notre objectif national de façon cohérente, avec l'ensemble des dimensions de l'aménagement du territoire. Ce volet du projet de loi est très technique, mais c'est la condition pour que ses dispositions soient opérationnelles. De fait, il y a encore de l'espace pour améliorer la clarté de certaines dispositions. Afin de préserver l'ambition écologique du texte, il est important pour le Gouvernement de redire quelles sont ses priorités. Il est essentiel d'avoir une définition claire et opérationnelle de l'artificialisation. Le Gouvernement présentera un amendement à l'article 48 visant à fonder la définition sur l'altération durable des sols et à préciser les modalités de décompte des objectifs dans les documents de planification. Il est également primordial de s'assurer que le dispositif proposé permette de territorialiser l'objectif d'une baisse de 50 % en tenant compte, monsieur le rapporteur pour avis, des disparités territoriales des grands projets qui peuvent intervenir, mais sans affaiblir notre ambition. Des améliorations peuvent encore être trouvées à la faveur de la navette parlementaire mixte paritaire. Nous portons aussi le rétablissement de la mesure de simplification de la mise en oeuvre des boni de constructibilité pour favoriser la densification ciblée en zone tendue, à l'article 51 A. concernant le sujet de l'urbanisme commercial, je redis clairement l'avancée majeure que représentent les articles 52 et 52 : l'interdiction stricte de tout nouveau centre commercial sur des terres agricoles ou naturelles de plus 10 000 mètres carrés et la mise en place d'un système de dérogations contraignant pour les surfaces de moins de 10 000 Je rappelle que le Gouvernement est extrêmement attentif au sujet des entrepôts de e-commerce, qui posent des questions d'équité fiscale, de mode de consommation et de modèle de société, mais aussi d'aménagement du territoire. C'est pourquoi la méthode que nous privilégions s'appuie, là encore, sur les territoires et la stratégie qu'ils déploient dans leurs documents de planification. Je ne doute pas que la qualité de nos débats à venir sur ces sujets essentiels pour les territoires et leur contribution à l'atténuation du changement climatique et à la résilience permettront d'avancer vers ces objectifs que nous partageons.

vise à exonérer des obligations relatives à la lutte contre l'artificialisation des terres les communes des territoires ruraux et, plus particulièrement, celles de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou encore constituée d'espaces naturels. naturels. Il serait contraire à l'esprit de la loi d'obliger ces communes à renoncer à des projets utiles pour leurs habitants et pour l'attractivité de leur territoire, alors qu'elles sont foncièrement ancrées en pleine nature et, partant, les plus respectueuses de l'environnement.

économiques ? Cet amendement vise à dispenser de l'application de la totalité de ce chapitre de loi relatif à l'artificialisation les petites communes rurales. Il cible les communes de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie est constituée d'espaces naturels ou agricoles.

n'a pas souhaité exclure purement et simplement ces communes du champ des dispositions sur lesquelles nous nous penchons aujourd'hui. D'abord, certaines dispositions de ce chapitre sont favorables aux communes, quelles qu'elles soient, notamment celles concernant la simplification ou les extensions des ORT. D'autres sont plus générales que la seule « zéro artificialisation nette », comme le moratoire sur les grandes surfaces. Ensuite, la grande majorité des petites communes rurales ciblées sont soumises au régime du règlement national d'urbanisme (RNU) : elles n'ont pas de document d'urbanisme et ne seront donc pas soumises aux objectifs chiffrés, au durcissement de certaines règles du PLU, aux obligations rédactionnelles. Enfin, la commission a modifié le texte tout au long de ce chapitre pour garantir la territorialisation et la différenciation, notamment en prenant en compte les enjeux ruraux ou la spécificité des communes déjà soumises à des restrictions foncières fortes. Nous allons poursuivre ce travail aujourd'hui. Vous le verrez, la commission sera favorable à plusieurs ajouts concernant le développement rural. Je pense que de nombreuses petites communes rurales de tradition agricole qui ont été confrontées ces dernières décennies à une urbanisation galopante partagent les objectifs et l'ambition de ce chapitre, notamment dans une optique de protection des terres agricoles. Pour toutes ces raisons, l'avis de la commission est défavorable. Quel est

Il prévoit deux objectifs distincts : d'une part, l'atteinte du « zéro artificialisation nette » en 2050, qui correspond à l'orientation fixée au niveau européen, et, d'autre part, une division par deux du rythme de l'artificialisation nouvelle sur une période de dix ans. En amont de nos débats, je souhaite dire un mot de cette logique de réduction de l'artificialisation nette, qui s'appliquera à l'échelle de la planification, c'est-à-dire des PLU et des SCoT. J'y insiste, il ne s'agit pas de dire que chaque particulier ou aménageur devra, pour chaque projet qui artificialise, acheter un terrain de même taille et le renaturer. Aucun projet individuel ne pourra être interdit sur cette base. Cela signifie, en revanche, que l'on regardera pour chaque PLU ou chaque SCoT, par exemple, le nombre d'hectares qui ont été artificialisés sur la période et le nombre d'hectares qui ont été désartificialisés : voilà ce qu'est l'artificialisation nette. Je proposerai tout à l'heure un amendement pour clarifier cette notion et sa définition, qui ont beaucoup occupé les débats de la commission. Je souhaite également rappeler que l'article 47 a une valeur programmatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement opposable au PLU ou au projet individuel, mais qu'il fixe simplement une orientation pour la Nation. En commission, nous avons souhaité réaffirmer, dès l'article 47, deux principes qui me paraissent fondamentaux : d'abord, ces objectifs sont fixés par la loi à une échelle qui est bien nationale ; ensuite, nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi que l'État garantira par les décrets ou les préfets l'application territorialisée et différenciée de ces objectifs, c'est-à-dire qu'il devra prendre en compte les spécificités locales et accueillir les projets de territoire des élus locaux. Plusieurs des amendements que nous allons examiner vont dans le même sens. Croyez bien que nous en partageons pleinement l'intention. C'est la raison pour laquelle, j'y insiste, notre commission a veillé à inscrire ces principes fondamentaux dès l'article 47.

« zéro artificialisation nette » ne doit pas brider ou annihiler les capacités d'accueil et de développement des communes rurales françaises. Il doit permettre de protéger- je pourrais dire sanctuariser -les terres agricoles nourricières. Sur ce point, la majorité de l'Assemblée nationale n'a pas pris ses responsabilités est restée dans une démarche d'imposition verticale définie par décret, échappant donc à tout débat démocratique, une fois de plus. En l'état, les maires, les élus locaux, ne pourraient à terme que constater les effets négatifs d'une procédure qui leur a complètement échappé, alors que le souhait de ruralité alimenté par le mal-être métropolitain n'a jamais été aussi présent. Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, ce n'est pas acceptable. Il ne suffit pas de s'affranchir de l'objectif pour que le problème disparaisse. C'est un point important du texte de la commission sur lequel nous sommes en désaccord, même si je tiens ici à saluer le travail du rapporteur pour avis Jean-Baptiste Blanc et du groupe de travail qu'il a piloté. Les démarches les plus efficaces résultent toujours de négociations entre parties prenantes. Imposer, on le sait, cela ne marche pas. Il faut, dans la négociation entre régions et communes ou EPCI, construire un calendrier réaliste qui nous permette d'être au rendez-vous de 2030 et de 2050. Il faut aussi savoir contractualiser le chemin à suivre et procéder ensuite à des évaluations régulières. C'est possible, mais pas avec le texte proposé. Nous vous présenterons un cadre de contractualisation avec la convention de sobriété foncière, qui doit indiquer le point zéro, l'état des lieux quantitatif de l'artificialisation et son évolution au cours des dix prochaines années.

Tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît. L'artificialisation augmente en effet presque quatre fois plus vite que la population. Les travaux de la commission ont abouti à réduire l'ambition de l'article d'atteindre » par « afin de tendre vers » l'objectif d'absence de toute artificialisation nette. Or, malgré un affichage de maîtrise de la consommation d'espaces depuis plus de trente ans, l'artificialisation des sols se poursuit. L'engagement national de réduction de l'artificialisation des sols est une mesure structurante pour l'avenir de nos territoires. Les objectifs doivent être affirmés clairement et sans ambiguïté. Notre amendement tend donc à revenir à la notion d'atteinte de l'objectif de ZAN pour 2050.

pour « tendre vers », en adoptant un amendement de notre collègue Stéphane Sautarel. Par cohérence avec cette position de la commission, je suis plutôt défavorable à ces amendements. Il ne nous semble pas opportun de continuer l'aller-retour entre ces deux notions et de revenir en arrière, d'autant que cette disposition

dans des ensembles urbains, soit inadaptées à des usages nouveaux. Nous avons donc besoin de la plus grande souplesse. Que les partisans du blocage de l'artificialisation le soient en pensant aux commerces

des moyens importants. De la même façon, sur le plan commercial, si vous voulez être certains qu'Amazon reprenne la totalité de la distribution dans notre pays,

Toutes les études démontrent que l'artificialisation fragilise la biodiversité en détruisant des habitats naturels ou en rompant la continuité écologique. Nous savons également qu'elle dégrade la capacité des sols à absorber l'eau, ce qui peut renforcer le ruissellement et aggraver les inondations. Les acteurs locaux sont conscients de ce défi. Mme Delattre, qui porte cet amendement,

ou des PLU intègre les problématiques de réduction de consommation de l'espace. L'urgence climatique impose une nouvelle étape, car si le plan de biodiversité de 2018 a posé le principe d'absence d'artificialisation nette à terme, celui-ci celui-ci n'a pas de valeur législative. Le présent article prévoit un double objectif de « zéro artificialisation nette » et une division par deux de l'artificialisation des sols en dix ans. Afin de sécuriser ces objectifs, l'amendement vise à retenir au sein de l'article 47 la notion de sobriété foncière, la notion d'artificialisation nette n'étant pas définie dans le code de l'urbanisme. de sobriété foncière, qui nous semble juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s'appuyer sur une notion d'artificialisation nette non définie dans le code de l'urbanisme pourrait ouvrir la porte à des contentieux portant sur des documents d'urbanisme. Quel est l'avis de économiques ? Je ne partage pas l'appréciation des auteurs de ces amendements, qui estiment que la notion de sobriété foncière est juridiquement et techniquement plus claire. Elle n'est pas définie par le droit ou par la pratique. Quels seront les indicateurs utilisés pour estimer si un document d'urbanisme est sobre foncièrement ou non ? C'est un vrai nid à contentieux, et je pense qu'il est préférable d'en préserver les collectivités locales- chacun en sera d'accord., notre commission a proposé une définition précise des sols artificialisés à l'article 48, pour compléter celle introduite par l'Assemblée nationale. Cette grille de lecture concrète est plus facile à prendre en main : elle permettra d'objectiver l'atteinte des objectifs. Il est donc plus sécurisant d'un point de vue juridique de se fonder sur la notion d'artificialisation nette que sur celle de sobriété foncière. Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements identiques. Quel est

entre des surfaces de terrains qui sont nouvellement artificialisés et celles de terrains renaturés et qui restaurent des sols agricoles naturels et forestiers. La sobriété foncière renvoie, elle, à un modèle d'aménagement durable qui vise à utiliser moins de terrain pour une fonction donnée. C'est l'un des leviers de lutte contre l'artificialisation des sols, mais ce n'est pas le seul. De plus, supprimer l'horizon temporel

celle-ci, c'est-à-dire de reculer l'échéance de cinq ans. Cette première étape nous paraît essentielle pour prendre en compte l'adaptation de cet objectif dans les différents documents de planification, mais également pour que les élus portent cet objectif dans le débat public et que les citoyens puissent se l'approprier. L'objectif ZAN implique en effet des changements importants de modèles de vie, voire des ruptures complètes qui requièrent l'adhésion des populations. Il convient donc de prendre en compte une phase de concertation avec les citoyens l'ensemble des acteurs, pour porter ce débat citoyen et favoriser ainsi l'acceptabilité et les réorientations induites par le ZAN. Il s'agit bien là d'une souplesse dans la mise en place et en aucun cas d'une remise en cause de l'objectif. économiques ? Cet amendement vise à reporter à 2035 l'atteinte de l'objectif de réduction par deux du rythme. Je partage, bien entendu, le constat des auteurs de l'amendement sur l'importance du débat public et du respect du cycle de vie des documents d'urbanisme. Nous avons d'ailleurs modifié en commission l'article 49, qui fixe les modalités de déclinaison dans les documents d'urbanisme afin de laisser davantage de temps pour intégrer les objectifs. La commission ne souhaite toutefois pas modifier la période de référence de dix ans, c'est-à-dire jusqu'en 2031. D'une part, elle permet d'avoir des données comparables sur la consommation d'espace sur une même durée, avant et après la loi. D'autre part, elle correspond aux échéances prévues par un bon nombre de SCoT. Je rappelle que presque 60 % des SCoT ont déjà inscrit une réduction de la consommation d'espace de 50 % ou plus. Je précise également qu'en commission nous avons apporté des modifications à l'article 49 qui permettront aux SCoT et aux PLU de fixer librement leur trajectoire de réduction. En conséquence, mon avis est défavorable. Quel est

économiques ? Je comprends tout à fait la crainte de voir les territoires qui ont consommé le plus d'espace bénéficier d'une forme de prime, tandis que ceux qui ont été les plus vertueux subiraient une forme de pénalité. Notre commission a été très attentive à ce que l'approche adoptée dans ce projet de loi ne soit pas punitive pour les collectivités qui ont été pionnières et volontaires. C'est la raison pour laquelle elle a adopté, à l'article 49, plusieurs amendements tendant à territorialiser l'application de l'objectif de ZAN en 2050, afin de tenir compte des spécificités et des trajectoires locales. Nous avons spécifiquement prévu que la déclinaison de l'objectif devra tenir compte des efforts de réduction de l'artificialisation déjà réalisés par les collectivités au cours des vingt dernières années. Il me semble que cela satisfait l'objectif de cet amendement et que cela permettra d'éviter cette prime aux moins vertueux. Par ailleurs, il ne me semble pas souhaitable de modifier la période de dix ans ; ce choix permet en effet de disposer de données comparables,

l'adaptation de la taxe d'aménagement ou par les abattements de plus-value immobilière. En matière de financement, le plan France Relance permet, au travers du fonds Friches, doté de 650 millions d'euros pour 2021-2022, de favoriser le portage d'opérations de recyclage des terres. Dans ce même cadre, une aide en faveur de la densification a été créée

Cet amendement a été déposé par nos collègues ultramarins. L'étude d'impact de ce projet de loi indique que, pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, « les données de l'observatoire national de l'artificialisation mettent en lumière une baisse significative du rythme de l'artificialisation. madame la ministre, qu'il convenait d'examiner ultérieurement le cas de ces territoires, chacun d'entre eux présentant des spécificités. Cet amendement a par conséquent pour objet d'acter dans la loi la définition d'une trajectoire sur mesure pour chacun de ces territoires.

de la commission des affaires économiques ? Les modalités de fixation des objectifs des collectivités et leur déclinaison territoriale ont constitué, tout au long de nos travaux, notre principal point d'attention. J'ai tenu à permettre davantage de différenciation locale et à rapprocher la décision de la réalité du terrain. Il est vrai que les collectivités d'outre-mer doivent faire face, à cet égard, à des problématiques particulières, liées à leur insularité et à la forte pression foncière qui y règne. Leur taux annuel d'artificialisation est relativement élevé en comparaison des autres territoires français, mais les enjeux de logement et d'aménagement ne sont pas comparables. Cela dit, la commission n'est pas favorable à une exemption des collectivités d'outre-mer des objectifs de limitation de l'artificialisation, pour deux raisons. raisons. D'une part, l'article 47 est programmatique ; il n'impose pas, en l'état, d'objectif chiffré spécifique à chaque territoire. La commission a d'ailleurs précisé que cet objectif programmatique s'applique bien à l'échelle nationale et ne sera pas opposable à chaque collectivité individuellement.

L'objectif pourra être fixé en fonction des enjeux locaux et il sera en effet possible de territorialiser, de définir localement, une trajectoire de réduction de l'artificialisation, en tenant compte des besoins spécifiques de ces territoires, par exemple en matière en matière de logement. La politique de lutte contre l'artificialisation reste un enjeu majeur pour ces territoires, qui disposent d'une biodiversité très riche et qui sont soumis à une forte croissance démographique. En outre, la réponse aux besoins de développement des territoires peut aussi se faire en optimisant l'utilisation du foncier, en particulier celui des espaces déjà artificialisés-

il convient de prendre en compte, à l'article 47, la spécificité des réalités locales en matière d'artificialisation des sols, en protégeant les capacités de développement

économiques ? En commission, sur l'initiative de nos collègues Anne Ventalon, Jean-Marc Boyer et Daniel Laurent, nous avons précisé que l'État devait garantir l'application différenciée et territorialisée des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols.

en matière de développement économique et démographique ou de préservation de l'activité agricole. Nous sommes tous confrontés, dans nos territoires, au départ des jeunes des zones rurales, faute d'habitat adéquat, d'emplois et de services. Nous savons que ces zones doivent être revitalisées, en opérant une mutation des bassins économiques, mais aussi en redynamisant l'activité agricole. L'enjeu est aussi celui de l'acceptabilité pour les élus de petites communes peu urbanisées, qui ne comprendraient pas que l'on sanctuarise leurs villages tandis que l'extension des grandes aires urbaines se poursuit. C'est pourquoi nous nous avons adopté en commission, à l'article 49, plusieurs amendements tendant à approfondir la territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation. Nous avons refusé une répartition des efforts décidée par la région au cours de grand-messes auxquelles les élus des communes ne seraient que peu associés. Nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi que les objectifs fixés dans les SCoT tiendront compte des besoins de revitalisation et de désenclavement rural et des enjeux spécifiques à la ruralité. En ce sens, l'amendement proposé est pleinement satisfait. Enfin- ce n'est sans doute pas délibéré -, la rédaction de cet amendement est en réalité plus restrictive que la rédaction actuelle, car elle conduirait à ce que l'État ne garantisse la territorialisation et la différenciation qu'aux zones rurales. Or c'est bien le développement pérenne et équilibré de chaque territoire, rural ou non, que nous entendons préserver. Pour toutes ces raisons, et au premier chef parce que nous considérons que l'intention des auteurs est pleinement satisfaite par l'article 49, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La parole est à M. le rapporteur pour avis. L'article 48 comporte deux grandes parties, qui font l'objet de très nombreux amendements. La première partie inscrit les objectifs de lutte contre l'artificialisation parmi les grands principes du code de l'urbanisme. La commission ne s'y est pas opposée ; elle est d'avis que l'artificialisation est, en effet, un grand enjeu de notre temps, qui doit être pris en compte par les politiques d'urbanisme et d'aménagement, à l'échelon local comme national. J'y insiste d'ailleurs, madame la ministre, l'État aménageur et constructeur doit s'astreindre à la même vertu que celle qu'il exige des des élus locaux et des collectivités. Au travers de ses amendements, notre commission a souhaité réaffirmer que la lutte contre l'artificialisation est, certes, une orientation forte, mais qu'elle n'est pas l'unique finalité de la politique d'urbanisme. Il ne faut pas penser en silos. Nous savons tous les injonctions contradictoires qui assaillent au quotidien les élus locaux : accélérer l'effort de construction de logements mais limiter l'étalement urbain ; développer les mobilités mais ne pas imperméabiliser ; relocaliser et réindustrialiser mais interdire les zones nouvelles d'activités économiques produire plus d'énergie renouvelable mais éviter les grands parcs photovoltaïques en zone agricole ; on pourrait continuer à l'infini ... En conséquence, la commission a souhaité équilibrer et articuler les objectifs existants du code de l'urbanisme, que je viens de citer, avec l'objectif relatif à l'artificialisation. C'est chose faite. C'est la raison pour laquelle nous ne serons pas favorables

place dans le code de l'urbanisme. Notre commission a donc souhaité que le Parlement se prononce sur une définition concrète, opérationnelle, afin que nous votions en toute connaissance de cause. Nous devons la clarté aux élus locaux ; si les documents d'urbanisme doivent être modifiés pour intégrer les objectifs chiffrés, il faut un classement et une comptabilité des sols artificialisés immédiatement mobilisables, transparents et surtout simples. Pas question pour les maires de devoir faire des études de sol aux quatre coins de la commune avant d'élaborer leur PLU ... Je me félicite de l'introduction en commission de cette définition complétée, qui nous paraît désormais opérationnelle et qui répond aux différentes attentes du terrain.

: La parole est à Mme Béatrice Gosselin. Il s'agit d'introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux. La lutte légitime contre l'artificialisation des sols ne doit pas empêcher les territoires ruraux et enclavés d'accéder au même niveau de développement que les territoires urbains et périurbains. En complément de l'objectif de zéro artificialisation nette, cette précision garantit l'égalité en droit de tous les citoyens.

aux territoires ruraux, qui font face à de multiples défis. Comme le proposent les auteurs de cet amendement, les grands objectifs du code de l'urbanisme mériteraient d'être complétés afin d'affirmer que l'urbanisme est non seulement au service des territoires urbains, mais encore au service du développement rural. Chaque territoire, quelles que soient ses caractéristiques,

le code prévoit déjà que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise le développement urbain maîtrisé. Ce principe général s'applique tant dans une commune urbaine que dans une commune rurale ; l'intention des auteurs de cet amendement est donc satisfaite. En d'autres termes, les enjeux majeurs de revitalisation des centres urbains mais aussi ruraux, d'équilibre des populations résidant respectivement en zones urbaines et en zones rurales, ainsi que de promotion d'un développement territorial lié aux besoins, sont déjà intégrés dans les objectifs assignés aux collectivités publiques agissant en matière d'urbanisme. l'article 48 a d'abord vocation à compléter ces objectifs généraux en y adjoignant les objectifs relatifs à la lutte contre l'artificialisation des sols, sans les opposer ni hiérarchiser, le présent projet de loi ne remettant pas en cause les objectifs existants. Néanmoins, j'ai bien conscience des enjeux de développement des territoires ruraux. C'est pourquoi le projet de loi prévoit une déclinaison, aux différentes échelles

intégré dans la stratégie de développement territorial de tous les projets publics et privés. Toutefois, cette ambition ne saurait être mise en oeuvre au détriment des territoires ruraux en perte démographique. doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensable à leur survie et au rééquilibrage des populations sur le territoire national. En outre, les communes rurales sont précisément celles dont la superficie de terrain artificialisé

Au risque de répéter ce qui a déjà été souligné, je rappelle que nombre de petites communes rurales situées en zone de revitalisation rurale ou ayant perdu des habitants au cours des vingt dernières années ne peuvent se permettre de limiter leur développement ; en outre, elles sont rarement les principales sources d'artificialisation des sols. La paralysie du développement rural demeure et constitue une donnée majeure et une préoccupation des élus locaux. Cette crainte est renforcée par l'application stricte des dispositions de la loi pour l'accès toute construction en dehors de l'enveloppe des villes-centres et des petits bourgs. Or, si les élus sont d'accord pour aller vers une certaine densification en réhabilitant autant que faire se peut l'existant, tout n'est pas réhabilitable. Il convient donc de permettre aux communes rurales de vivre et de se développer pour accueillir de nouveaux habitants ainsi que les services nécessaires à leurs besoins. Le potentiel de développement des petites communes rurales n'a, en effet, pas besoin d'être davantage contraint qu'il ne l'est déjà. Le désengagement de l'État, la destruction des services publics, particulièrement de leurs antennes dans nos territoires ruraux, et la désertification médicale et scolaire qui les touchent suffisent à leurs difficultés. Cet amendement vise donc à prévoir que la politique de lutte contre l'artificialisation des sols tienne compte des disparités de développement sur le territoire et équilibre les efforts fournis, selon une péréquation prenant en considération les besoins de développement des communes. Varaillas. Les motivations sont les mêmes ; cet amendement vise à affirmer la prise en compte de la situation particulière des communes rurales les plus fragiles démographiquement,

mais les communes très peu denses.

Vouloir repenser l'urbain sans prendre en compte le potentiel offert par le rural accentuerait les ruptures territoriales ; je rappelle qu'un tiers de la population vit dans une commune rurale, selon la dernière étude de l'Insee sur. C'est bien une profonde évolution de notre rapport à la ville et aux territoires qu'il faut engager, dans un objectif de préservation et de cohésion. Notre amendement tend ainsi à intégrer, dans la liste des équilibres à trouver pour mettre en oeuvre l'objectif de ZAN, la prise en compte des enjeux propres aux territoires ruraux.

cet amendement ; il s'agit de donner suite aux différentes demandes exprimées lors des débats parlementaires et aux échanges intervenus avec les associations nationales de collectivités. Ces échanges ont révélé la nécessité de préciser encore la définition de l'artificialisation

L'amendement du Gouvernement tend donc à distinguer le processus d'artificialisation qui résulte d'une altération durable des fonctions d'un sol par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux. Cette définition tient compte du degré d'atteinte aux fonctionnalités des sols et ne se limite pas à la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. L'objectif de zéro artificialisation nette fait l'objet d'une considération distincte dans les documents de planification et d'urbanisme. Il s'entend comme l'équilibre bilanciel entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées. tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l'objectif de limitation de l'étalement urbain et du mitage en dehors des zones urbanisées avec celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques dans les zones urbanisées. Dans un second temps, le décret permettra de détailler les modalités d'application de cette disposition et, plus particulièrement, le décompte à la parcelle à l'échelle des PLU et des cartes communales. : La parole est à M. Daniel Salmon. L'amendement du Gouvernement vise à définir l'artificialisation des sols par une altération durable des fonctions d'un sol entraînée par un projet de construction, d'aménagement, d'installations ou de travaux. Cette définition tend à rétrécir le champ de l'artificialisation, car d'autres facteurs, autres que des projets de construction,

de différencier entre artificialisation d'extension et artificialisation dans l'enveloppe urbaine existante. Cet amendement vise à affiner cette définition. Il est en effet impossible de mettre à égalité, en matière d'artificialisation, l'extension des zones urbaines, qui grignote les terres agricoles, les forêts et les espaces naturels, et l'artificialisation qui a lieu au sein d'aires urbaines déjà comparativement pauvres en biodiversité. Alors que 596 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés en dix ans, il est urgent de mettre un frein à l'extension des aires urbaines. De plus, en nous appuyant sur la notion d'« espace agricole, naturel ou forestier », nous proposons d'harmoniser la définition des espaces non artificialisés avec celle qui est déjà utilisée par les services déconcentrés de l'État comme les la définition du critère d'imperméabilisation permet également d'insérer une dimension qualitative mesurable dans l'article. Ces deux éléments permettent ainsi d'opérationnaliser la définition de l'artificialisation des sols et d'en faire un outil de politique publique efficace. Les trois amendements suivants sont

ainsi que son potentiel agronomique. Le présent amendement vise à fonder cette définition sur la réduction des espaces agricoles, naturels ou forestiers, conformément à l'objectif fixé par la loi, et à y intégrer un objectif qualitatif relatif à la réduction de l'imperméabilisation. Ces deux notions sont maîtrisées par les élus locaux et sont gages d'une meilleure mise en oeuvre du dispositif. La parole est

écologiques du sol, risque d'obérer le déploiement des énergies renouvelables. Or celles-ci peuvent se développer en préservant, voire en améliorant la biodiversité locale, l'imperméabilisation des sols étant négligeable à l'échelle des parcelles, et surtout en

l'énergie photovoltaïque, l'installation des panneaux photovoltaïques répond à une directive qui impose aux entreprises d'organiser la collecte et le traitement des équipements usagés. La définition de l'artificialisation doit donc intégrer le nécessaire déploiement des énergies renouvelables en tenant compte de leurs propriétés vertueuses en matière de préservation de la biodiversité et de transparence hydraulique.

Afin de rendre la portée de la définition de l'artificialisation des sols au sein des PLU plus ambitieuse et plus claire, il est proposé de remplacer le mot « principalement » par le mot « majoritairement ». Serait donc considéré comme artificialisé un sol dont au moins 50 % de la surface serait imperméabilisée.

par un paragraphe censé expliciter la notion d'artificialisation. À mon sens, cet amendement n'est pas du tout source de clarté. Il y est fait référence à des notions toujours très vagues, comme « [l]es surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ». De surcroît,

si le sol est restauré et si la zone est transformée en forêt, ledit terrain pourra être considéré comme désartificialisé. Si l'on ne comptabilise que les atteintes qui tuent pour toujours un sol, une grande partie de l'artificialisation sera donc invisible. Enfin, l'amendement

dans l'amendement du Gouvernement peuvent altérer durablement les fonctions du sol. Le Gouvernement estime, au contraire, que cette formulation permet de couvrir toutes les actions d'aménagement et d'urbanisation visées par la réforme. Cette rédaction est également conforme à la nomenclature des catégories de projets soumis à évaluation environnementale. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ce sous-amendement,

présenter l'amendement n° 660 rectifié. Si des actions volontaires en matière de lutte contre la consommation des sols et des espaces naturels doivent être entreprises pour répondre à l'enjeu de protection de la biodiversité, il convient également de prendre en compte les autres politiques pour lesquelles il est également demandé d'accentuer les efforts. La commission a d'ailleurs modifié l'article 48 afin que l'objectif de limitation de l'artificialisation des sols n'omette pas la nécessité de concilier la maîtrise de l'étalement urbain avec l'ensemble des objectifs en matière d'habitat, de prévention des risques, de mobilité ou de ruralité. C'est une bonne chose. Dans cet esprit, l'amendement de Mme Delattre vise à supprimer, dans la définition de l'artificialisation, la mention selon laquelle « les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées », afin de ne pas entraver la densification des zones déjà bâties. La parole est à M. Daniel Salmon, l'amendement n° 912. Cet amendement tend à exclure, dans la définition de l'artificialisation adoptée par la commission, les surfaces de pleine terre des sols non artificialisés. Les débats à l'Assemblée nationale ont conduit à introduire cette notion pour en faire un levier contre l'artificialisation en ville. La préservation de la pleine terre peut en effet constituer un outil de lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain et contre les risques d'inondation par ruissellement. notamment les PLU, y font de plus en plus fréquemment référence, mais chacun a le plus souvent sa propre définition. En effet, la notion de pleine terre n'est pas définie ; il est donc risqué d'associer cette notion, encore floue juridiquement, à la définition de l'artificialisation, sujet on ne peut plus complexe où chaque mot pèse.

parole est à Mme Micheline Jacques. L'objet de cet amendement est de permettre le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain

Cette obligation est actée préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter. Des garanties financières prises par l'exploitant permettent de surcroît à l'administration de pallier immédiatement une éventuelle défaillance. Bien souvent, cette action contribue à développer ou à préserver la biodiversité de ces espaces restitués. Ainsi, il semble qu'intégrer les carrières aux terrains artificialisés ne tiendrait pas compte de la réalité de ce secteur

visait à clarifier le sort des terres agricoles ou encore de certains espaces comme les jardins et les parcs. La commission s'était donc opposée à sa suppression. Toutefois, la définition que nous avons adoptée en commission précise désormais explicitement que les terres à usage de culture et les zones végétalisées attenantes au bâti ne sont pas artificialisées. La phrase relative à la pleine terre, moins précise juridiquement, est donc désormais superflue.

de réhabilitation assorties de garanties financières, je comprends l'intention de son auteur mais la commission y est défavorable. Même si une renaturation est prévue à terme par la loi, le sol n'en est pas moins artificialisé durant la période de l'exploitation,

Il ne nous semble pas opportun d'exclure si précisément ce seul type d'installation photovoltaïque, alors que le but de l'inscription de la définition à ce niveau du code de l'urbanisme est de lui donner

peuvent porter atteinte au sol de façon durable. Il n'est donc pas opportun de prévoir ainsi une telle exclusion dont les effets affaibliraient considérablement la portée de la réforme ambitieuse prévue par le présent projet de loi.

proposée à l'alinéa 9 de l'article 48 est trop large et trop floue. Elle peut conduire à considérer que certaines pratiques agricoles- drainage, irrigation, apport d'amendements, utilisation de produits phytosanitaires -affectent l'usage des sols agricoles et les font basculer dans la catégorie des sols artificialisés. Or l'objectif premier de ce volet du projet de loi est de lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation. Pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation future de la définition des sols artificialisés et ainsi limiter les contentieux, il est proposé d'ajouter à la définition existante que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier

Je suis tout à fait en phase avec l'intention des auteurs de cet amendement. D'ailleurs, la rédaction adoptée par notre commission, qui propose une nouvelle définition, plus opérationnelle, de l'artificialisation, précise que les surfaces nues, c'est-à-dire naturelles, à usage de cultures- agricoles ou sylvicoles -ainsi que la plupart des surfaces végétalisées ne sont pas artificialisées. Votre intention est donc satisfaite,

Cet amendement vise à préciser que les friches et délaissés urbains sont considérés comme artificialisés, afin que les projets réalisés sur ceux-ci ne soient pas pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation.

qui sont des zones inutilisées nécessitant une réhabilitation. Si les friches sont considérées, au début de la période de référence, comme étant déjà artificialisées, les constructions réalisées sur ces friches, qui contribueront au recyclage foncier, ne seront pas comptabilisées comme de l'artificialisation nouvelle.

du Gouvernement ? Nous considérons qu'il n'est pas opportun que la loi procède à une catégorisation fine des surfaces artificialisées ou non artificialisées en ne ciblant que certains secteurs ou types d'occupation, d'usage ou de terrain. Le décret en Conseil d'État fixera une nomenclature répondant à cet objectif. J'ajoute que les friches agricoles, par exemple, sont potentiellement non artificialisées,

économiques ? Cet amendement vise à renforcer les conditions d'ouverture à l'urbanisation. Il est prévu que de telles ouvertures ne peuvent intervenir que si les projets ne peuvent pas être réalisés sur des espaces déjà artificialisés.

que les PLU et les cartes communales ne peuvent rendre de nouveaux secteurs constructibles qu'en justifiant « que la capacité de construire ou d'aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés » et même, pour les PLU, en réalisant une autre étude de densification. L'intention des auteurs de cet amendement me paraît donc pleinement satisfaite. Avis défavorable. Quel est

la commission des affaires économiques ? L'objet de cet amendement est que l'impact des grands projets d'envergure nationale ou régionale ne soit pas pris en compte dans l'évaluation des objectifs de lutte contre l'artificialisation. Je partage absolument cette intention. Il est souhaitable que ces projets, qui bénéficient à tout un territoire, ne pénalisent pas les communes qui les portent. Je pense à des gares TGV, à des opérations d'aménagement structurantes, à des installations portuaires et à tant d'autres cas.

du Gouvernement ? L'adoption de cet amendement ainsi rédigé conduirait à exclure un grand nombre de constructions, d'aménagements, d'équipements et d'infrastructures pouvant entraîner une artificialisation des sols.

permettent en effet un fonctionnement optimal de l'organisation territoriale du point de vue de l'accès des habitants aux équipements et aux services. L'action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en matière d'accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l'enseignement ou encore les transports. Afin de ne pas pénaliser ces communes-centres, sièges de services et de fonctions à caractère urbain, il est proposé que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée. Quel est l'avis de

ou de prise en compte du Sraddet le permet tout à fait. Si c'est l'EPCI qui est compétent en matière d'urbanisme, alors l'objectif de réduction de l'artificialisation est de toute façon déjà mutualisé à l'échelon intercommunal. Il n'est donc pas besoin de le pondérer. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, hydriques et climatiques, dont le fait qu'elles soient affectées conduit à considérer la surface comme artificialisée, l'objectif étant de prendre en compte le degré d'atteinte aux différentes fonctions des sols. Cette approche implique une profonde transformation des pratiques. Il y a en effet un fort enjeu à ce que les outils de suivi soient en phase avec la définition retenue et ne se réduisent pas à un simple suivi surfacique de la consommation d'espace. L'article 48 renvoie à un décret le soin d'établir une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, et de déterminer l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée. Nous proposons que ce décret fixe également les indicateurs qui permettront de caractériser les fonctions du sol avant son artificialisation et d'apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

J'avoue avoir des doutes quant à sa portée concrète. En effet, les travaux de la commission des affaires économiques ont mis en avant une triple nécessité : d'abord, offrir aux élus locaux un dispositif aussi concret et opérationnel que possible, ensuite, sécuriser les documents d'urbanisme et les décisions des communes face aux risques de contentieux que nous avons évoqués à plusieurs reprises, enfin, éviter d'alourdir les procédures et les charges nouvelles qui incomberont aux collectivités. La définition et la nomenclature prévues par cet article visent justement à créer un nombre fixe de catégories de sols artificialisés et non artificialisés qui soient directement mobilisables par les communes et les EPCI et qui puissent être intégrées

Notre objectif est d'éviter d'associer deux statuts différents à un même sol au regard de son admissibilité à être cultivé et de son artificialisation. Il s'agit donc de faciliter l'application du présent texte, en particulier pour les territoires à forte composante agricole. Quel est l'avis de

Il a pour objet d'inscrire la priorité d'utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement. La préservation de nos forêts est un enjeu majeur pour lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. La Convention citoyenne pour le climat a proposé d'encadrer strictement les coupes rases, de renforcer les effectifs de l'Office national des forêts (ONF) ou encore de faire évoluer le code forestier pour mieux intégrer les enjeux écologiques. Cet amendement vise à répondre à l'une de ces attentes en inscrivant au sein du code forestier l'encadrement des autorisations de défrichement, tout en participant à la lutte contre l'artificialisation des sols que promeut l'article 48. Cette rédaction Cette rédaction est inspirée de l'article 5 de la loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, lequel est encore plus restrictif, puisqu'il impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé qu'à l'endroit prévu. Quel économiques ? Cet amendement vise à renforcer la conditionnalité de la délivrance de l'autorisation de défrichement des surfaces boisées, en n'autorisant le défrichement que lorsque le projet envisagé ne peut pas être réalisé sur des sols déjà artificialisés. Cette discussion prolonge en réalité nos débats relatifs à la maîtrise de l'urbanisation et à la protection des espaces forestiers. La rédaction proposée n'empêche pas le défrichement lorsque celui-ci est justifié par la nécessité et compensé comme le prévoit la loi, mais elle offre une garantie supplémentaire pour la protection des bois et des forêts. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement. du Gouvernement ? L'autorisation de défrichement n'a pas vocation à autoriser un projet, mais elle peut refuser le défrichement nécessaire à la réalisation du projet sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt de celui-ci. En effet, le Conseil d'État s'est prononcé sur les autorisations de défrichement et a affirmé que le défrichement devait être apprécié sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises. ailleurs, la lutte contre l'artificialisation permet déjà de tenir compte de la préservation des espaces forestiers, plus particulièrement des sols forestiers. C'est en effet l'un des enjeux pris en compte pour l'atteinte de l'objectif d'absence de toute artificialisation nette mentionné à l'article 48. L'approche défendue dans ce projet de loi est celle d'une réduction de l'artificialisation organisée par les collectivités dans leur exercice de planification. Ainsi, l'implantation d'un projet sur un espace nécessitant un défrichement ne sera possible que si le document d'urbanisme l'autorise, au regard des objectifs du présent projet de loi, à savoir une ouverture à l'urbanisation justifiée par l'impossibilité de répondre aux besoins dans les espaces urbanisés et conforme à la trajectoire de réduction de l'artificialisation fixée par le document.

Martin Lévrier. Cet amendement déposé par Julien Bargeton vise à prendre en compte le développement du télétravail parmi les objectifs de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Concrètement, cette consécration pourrait aider, en cas de contradiction avec d'autres objectifs, à la réalisation de projets tels que la construction de télécentres ou de travaux accessoires comme le raccordement de vieux bâtiments désaffectés à des réseaux nécessaires au fonctionnement des tiers-lieux.

En ce sens, cet amendement est satisfait. D'autre part, il semble préférable de conserver à cet article son caractère général, c'est-à-dire un recensement d'objectifs principaux, sans trop entrer dans le détail. En y faisant figurer expressément le télétravail, nous entrons dans un degré de précision qui ne correspond pas à l'ambition de l'article plus les objectifs sont précis, moins leur conciliation est aisée. En tout état de cause, l'essor du télétravail trouverait davantage sa place dans le code du travail que dans le code de l'urbanisme. Avis défavorable. du Gouvernement ? L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme fixe les objectifs généraux que doit viser l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, notamment au travers de leurs documents d'urbanisme. L'accès à des locaux dédiés au télétravail, s'il est nécessaire, peut déjà s'inscrire dans les objectifs de diversité des fonctions urbaines, qui doivent inclure la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques et d'équipements publics, en tenant compte notamment des objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'accès à de tels locaux relève de l'usage des bâtiments, donc pas du champ de la loi ni de celui des documents d'urbanisme ; ces derniers peuvent réglementer la destination des sols et des constructions, en visant la mixité des fonctions urbaines, mais n'ont pas à intervenir sur leurs différents usages. Il me semble donc nécessaire

n° 957 rectifié. La commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol,

compléter le code de l'environnement par un article additionnel portant définition des sols et des sous-sols afin de caractériser leurs fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles et, bien entendu, de les sanctuariser.

les sols ne sont pas traités par le code de l'environnement en tant que ressource naturelle à protéger face aux changements climatiques et aux dégradations. Des travaux avaient été engagés à l'échelon européen pour élaborer une grande directive-cadre sur la protection des sols, mais ils sont au point mort depuis de nombreuses années.

à cette proposition ambitieuse par laquelle la France pourra être le fer de lance de l'effort de protection des sols. La rédaction proposée vise le code de l'environnement. Elle complète utilement la définition des sols artificialisés et non artificialisés introduite dans le code de l'urbanisme par le projet de loi. Elle détaille notamment les fonctions des sols.

leur exclusion poserait de nombreux problèmes quant à la portée des opérations de dépollution. Par ailleurs, la volonté de protéger le sol et le sous-sol contre les processus naturels soulève de nombreuses questions en matière de priorisation de l'action de l'État. Enfin, les définitions proposées

et de gestion de l'eau, à l'élaboration des SCoT. Toutefois, la rédaction initialement proposée avait aussi pour effet de prévoir une association systématique de ces établissements publics à l'élaboration ou à la révision de tous les PLU. que je vous soumets est plus fidèle à l'intention première, qui est de mieux intégrer les enjeux de gestion au SCoT, échelon pertinent, sans alourdir les procédures relatives au PLU. En outre, le PLU doit déjà respecter les prescriptions du SCoT en matière de « trame bleue » et de traduction du schéma